Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l'examen de l'article 1.

pour une raison très simple, que notre collègue vient d'expliquer : le rapport de subordination des salariés envers les employeurs. Quiconque a déjà été salarié ou employeur sait pertinemment qu'il y a un rapport de domination de l'un sur l'autre. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'ont émergé les organisations syndicales qui, par leurs droits collectifs d'expression et d'action, peuvent pour partie rétablir l'équilibre des rapports de force dans une négociation. L'alinéa 12 permet à un employeur d'organiser la signature d'un accord sans les organisations syndicales, mais par le biais d'élus du personnel sans mandat syndical. Il remet en cause ce principe de négociations peu ou prou équilibrées. Vous le savez, les syndicats se forment pour connaître les textes qui régissent le droit du travail et ce n'est pas le cas pour des personnels sans appartenance syndicale. Ainsi, des salariés sans appui syndical, potentiellement soumis à des pressions patronales sur l'emploi, pourront négocier des accords au risque de se faire imposer des décisions contraires à leur intérêt. Vous ne faites donc que renforcer le pouvoir de domination de l'employeur sur l'employé en permettant le contournement des organisations syndicales qui sont pourtant les garantes d'une force collective de négociation. Finalement, la mesure proposée à l'alinéa 12 de cet article permet la généralisation du chantage à l'emploi et l'affaiblissement des droits collectifs d'organisation des salariés. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, mes chers

95 visent à supprimer l'alinéa 12, donc les apports de la commission. Je rappelle une évidence : personne ne peut obliger un salarié à devenir délégué syndical ou à être mandaté. Or, comme la conclusion d'un accord est aujourd'hui par principe un monopole du délégué syndical, les petites entreprises et leurs salariés se retrouvent à l'écart de la négociation collective. Doit-on accepter cette situation ? accepter cette situation ? Doit-on fermer les yeux et ne s'occuper que des entreprises dotées de délégués syndicaux ? La réponse est évidemment non. C'est pourquoi nous avons voulu trouver une solution pragmatique pour encourager le dialogue social dans les petites entreprises sans délégué syndical.

qui adhèrent à un syndicat, sont élus au premier tour des élections de délégués du personnel, mais ne veulent pas être délégués syndicaux. C'est une réalité quotidienne. Les délégués du personnel me paraissent tout à fait aptes à négocier. Le dernier cas est celui de la consultation

nous proposons cette fois-ci de supprimer l'habilitation donnée au Gouvernement de faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord. Certes, la formulation « consultation des salariés [ ...] pour valider un accord » pourrait paraître positive et représenter un véritable signe de dialogue social tel que nous le concevons, mais, en y regardant de plus près, la dimension de cette consultation est quelque peu particulière, pour ne pas dire partisane. En effet, l'objectif réel de cette disposition est de contourner les syndicats. Bien évidemment, pour qu'un accord dérogatoire d'entreprise soit valable, il faut qu'il soit adopté. La loi El Khomri a déjà permis

que ce référendum à l'initiative de l'employeur est une grande revendication du MEDEF. Cela n'est pas pour nous étonner et, si certains se faisaient des illusions sur le but du Gouvernement ou sur la proximité de vue entre le Président de la République et les organisations patronales, ils trouveront ici une preuve concrète de leur naïveté Derrière un argument démocratique et populaire- le référendum -, c'est l'existence et la légitimité mêmes des syndicats représentatifs qui sont attaquées. Finalement, on pourrait faire une analogie entre ce référendum à l'initiative de l'employeur visant à dire aux syndicats « circulez, il n'y a rien à voir » et ces ordonnances qui disent la même chose aux parlementaires, tout cela bien sûr sous couvert de dialogue social et de modernité. Les pouvoirs jupitériens du Président de la République s'accompagnent de pouvoirs tout aussi jupitériens des employeurs. Dans les deux cas, les représentants du peuple, des collectivités ou des salariés sont contournés, et ce, nous n'en doutons pas, dans l'intérêt du plus fort ! Pour résumer, cet alinéa 13, qui se pare d'une belle apparence démocratique, constitue un véritable danger et un chèque en blanc donné aux employeurs, c'est pourquoi nous en demandons la suppression. L'amendement n° Ce projet de loi élargit tant le champ de la primauté de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche que les possibilités de négociation en l'absence de délégué syndical. Dans ce cadre, l'alinéa 13 de cet article propose de favoriser les conditions de mise en oeuvre de la négociation collective en « facilitant le recours à la consultation des salariés, notamment à l'initiative de l'employeur, pour valider un accord ». À l'image de l'ensemble du texte qui nous est soumis, cette proposition nous semble pour le moins floue. Selon nous, toute consultation devrait au minimum respecter règles. Tout d'abord, en matière d'information : les tenants et les aboutissants de l'accord doivent être notifiés clairement et de manière intelligible. Ensuite, le périmètre de cette consultation doit être raisonnable et réfléchi. En effet, pour qu'une consultation soit juste, elle doit faire appel à l'avis des employés mêmes qu'elle concerne. Si un accord impose, par exemple, le travail de nuit aux ouvriers d'une entreprise, les cadres de cette même entreprise non concernés par la mesure ne peuvent être invités à s'exprimer sur cet accord. Cela relève du bon sens, mais mérite d'être précisé, afin d'éviter tout détournement du processus.

s'agit de maintenir la présence syndicale au sein des petites entreprises. La commission des affaires sociales a souhaité permettre à l'employeur d'organiser un référendum pour valider un projet d'accord afin de surmonter l'opposition des syndicats majoritaires.

Cet amendement vise un sujet dont nous avons eu l'occasion de débattre l'an dernier. En effet, depuis la loi El Khomri, un accord peut être validé par seulement 30 % des organisations syndicales

Cela paraît d'autant plus regrettable que le Gouvernement doit rendre au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application des nouvelles règles de majorité relatives aux accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés, ainsi qu'aux accords de préservation ou de développement de l'emploi. Sans attendre, on légifère à nouveau ! Une méthode permettant de renforcer le dialogue social consisterait à attendre ce rapport, ce qui nous permettrait d'évaluer utilement l'opportunité de généraliser, par un acte législatif, de nouvelles règles de validité pour l'ensemble des accords collectifs. En effet, il faut le rappeler, le risque de court-circuiter les organisations syndicales existe, des exemples récents ayant montré que le recours au référendum d'entreprise est trop souvent utilisé comme un outil de contournement des syndicats. S'il existe des blocages, ce n'est pas par défiance envers le dirigeant d'entreprise, mais parce que les solutions proposées ne conviennent pas à plus de 50 % des salariés et à plus de 30 % des organisations syndicales. Ce sont bien ces seuils qui garantissent que les syndicats représentants et élus du personnel peuvent jouer leur rôle au sein de l'entreprise. Ils apportent une garantie au maintien des corps intermédiaires dont, pourtant, l'article 2 du présent texte loue

n 27 rectifié et 96, contrairement à ce que pensent nombre de nos collègues, il est déjà possible pour un employeur d'organiser un référendum en vue d'entériner un accord, par exemple en matière d'intéressement

Le Gouvernement a la volonté de développer les référendums décisionnels. Nous partageons cette ambition et avons seulement rappelé que ces référendums doivent aussi pouvoir être déclenchés par l'employeur et non seulement par les syndicats, par parallélisme des formes.

je crois qu'il ne faut pas, mon cher collègue, être méfiant à l'excès à l'égard des outils de démocratie directe, qu'il s'agisse de la démocratie politique ou de la démocratie sociale. Vouloir développer un peu le référendum décisionnel dans les entreprises n'est pas incompatible avec le dialogue avec les syndicats. Le dialogue social peut avoir plusieurs facettes, sans créer de monopoles d'aucune sorte. amendement vise à encadrer, plutôt qu'à faciliter, le développement des consultations des salariés. Les auteurs de cet amendement sont donc à l'opposé de la philosophie du Gouvernement et de la commission sur ce point, c'est pourquoi celle-ci a émis un avis défavorable sur cet amendement. L'amendement n° L'amendement n° 191 n'est pas acceptable, car il tend précisément à revenir sur les travaux de la commission des affaires sociales. Je tiens à préciser un point : la commission et moi-même sommes opposés à la généralisation des accords majoritaires, mais si celle-ci doit être maintenue, il convient de donner à l'employeur, et non seulement aux syndicats minoritaires, la possibilité d'organiser un référendum pour faire valider un accord. C'est une question d'équité entre employeur et syndicats dans l'entreprise.

dans la loi d'habilitation, à l'article L. 2232-12 du code du travail, qui consacre justement cet accord majoritaire, généralisé à partir de 2019. Ce serait envoyer un signal contradictoire de la part du Sénat. La commission a donc émis un avis défavorable. Quel est

dans le respect, bien sûr, des règles fixées par l'OIT et par la convention de Genève. C'est ce calibrage fin que nous sommes en train de ciseler avec les partenaires sociaux. Encore une fois, il ne s'agit pas d'en faire un outil permanent

ont voté contre, mais que le périmètre de ce référendum incluait des cadres qui, eux, ont voté pour. Finalement,

faire preuve de méfiance vis-à-vis du dialogue social que de demander que les référendums soient encadrés ; les points que j'ai soulevés dans mon intervention visaient précisément cet exemple.

de certaines avancées réalisées par les organisations syndicales et qui vont plutôt dans le sens d'une conciliation avec l'autre partenaire social. Si vous ne l'acceptez pas, mes chers

À l'Assemblée nationale, vous avez rappelé que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel seraient saisis. Or le Conseil constitutionnel ne vérifiera pas que la comptabilité entre les lois d'habilitation et de validation et le texte de l'ordonnance ! Vous devrez saisir le Conseil d'État, mais celui-ci ne rendra qu'un avis et, une fois la validation votée, il ne pourra plus juger des mesures qui se trouvent dans l'ordonnance, la loi faisant écran. Cette commission remodelée aurait pu apporter des garanties supplémentaires, dont cet alinéa nous prive. C'est d'autant plus regrettable que la vocation de votre réforme est de changer en profondeur un droit qui est essentiel à la vie des salariés.

nous assure qu'il sera en mesure de publier rapidement l'ordonnance pour clarifier l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise et remplir ainsi les objectifs de la feuille de route fixée par la commission de refondation. de refondation. J'avoue avoir été longtemps perplexe, madame la ministre, car le rapport Combrexelle prévoyait qu'il faudrait quatre ans pour refondre le code du travail.

de refondation est rendue sans objet par la loi et les ordonnances qui seront prises sur son fondement. En effet, le but de cette commission était d'attribuer une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et de son champ d'action, et de réécrire, sur cette base, toute la partie du code du travail concernée.

peu déçu d'avoir eu raison lorsque nous avons montré à Mme El Khomri qu'elle mettait la dynamite dans le code du travail et qu'il suffisait qu'un nouveau gouvernement entre

y compris par les parlementaires.

à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun lien de subordination entre le franchiseur et les salariés des franchisés. Les franchisés disposent eux-mêmes

à l'article 38 de la Constitution, qui interdit aux amendements parlementaires de créer une habilitation à légiférer par ordonnance. Je partage néanmoins le souci de notre collègue Jean-Marc Gabouty de supprimer cette instance, conformément à la position exprimée

Cet amendement vise à revaloriser le SMIC brut à 1 800 euros à compter du 1 janvier 2018, soit un peu moins de 1 400 euros nets mensuels. Un quart des Français gagnent moins que cette

une dizaine d'années, la hausse annuelle moyenne a été d'environ dix centimes ? Cependant, les rémunérations moyennes des responsables exécutifs des entreprises du CAC 40 sont passées, elles, de plus de 3 millions d'euros à presque 5 millions en 2015, soit une hausse de 63 % en six ans. La quasi-stagnation des salaires limite la demande, donc la production de biens manufacturés et de services. Ce mécanisme entretient en fait une spirale déflationniste, une course aux prix bas dangereuse pour les emplois, les conditions de travail et l'environnement. C'est pourquoi il nous semble que la question de la rémunération du travail doit être au coeur de nos travaux, travaux, sur ce texte comme sur d'autres. Tel est le sens de cet amendement d'appel. Mme la ministre a dit hier qu'il fallait s'attaquer à tous les problèmes en même temps. Les très bas salaires en sont un ! Quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet ?

de certains travailleurs entraîne comme effet pervers des trappes à pauvreté. Certaines personnes restent au chômage, car leur productivité n'est plus suffisante pour un salaire donné. Conservons les règles actuelles d'indexation du SMIC pour l'instant.

ce point est hors champ du projet de loi, je souhaite rappeler que les mécanismes de revalorisation existent dans le code du travail. Ils sont prévus après consultation des organisations syndicales et professionnelles. Je ne puis donc qu'être défavorable à cet amendement. Ce n'est pas le bon lieu ni la bonne méthode.

secteur des services, où il y a peu de concurrence, que les bas salaires pèsent le plus. Nous avons besoin, pour la relance de notre économie, pour les carnets de commandes de nos entreprises, d'avoir une juste rémunération

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

scrutin est ouvert.

d'une prime. Ce périmètre bien trop large de la définition du licenciement économique a fait l'objet de fortes contestations lors des débats sur la loi El Khomri. Nous profitons du débat de ce soir pour demander l'abrogation

: La parole est à Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à réintroduire la validation obligatoire de la commission de validation des accords collectifs pour les accords conclus par des élus non mandatés. Cela permettra de répondre à une double inquiétude exprimée lors de la présentation de notre amendement de suppression, à savoir, d'une part, le renforcement du rôle régulateur de la branche et, d'autre part, la remontée effective des informations de terrain au niveau de la branche.

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à supprimer une souplesse procédurale introduite par la loi Travail. En outre, je souhaite une refonte globale des règles de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, comme y invite l'alinéa 12 de l'article 1 tel que réécrit par la commission. L'article L. 2232-22 du code du travail prévoit actuellement que les accords conclus par des élus du personnel non mandatés doivent seulement être transmis pour information à la commission paritaire de branche. L'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur des accords. Le Sénat plaidait depuis 2015 pour cet assouplissement, car toutes les branches n'ont pas mis en place cette commission paritaire. Et lorsqu'elles existent, ces commissions tardent à rendre leur décision, voire exercent un contrôle d'opportunité et non de légalité des accords. L'alinéa 12 de l'article 1, que nous venons d'adopter, doit lancer le chantier d'une refonte des règles de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. On ne peut, d'un côté, donner au Gouvernement une habilitation et, de l'autre, traiter directement ce sujet dans le code du travail.

Au travers de cet amendement, nous souhaitons supprimer une disposition introduite par la première loi Travail dans ses articles 16 et 21. En effet, l'article L. 2242-20 du code du travail, issu des débats de l'été dernier, permet l'adaptation des règles de négociation par voie d'accord d'entreprise et ainsi de déroger au droit commun défini par l'article L. 2242-1 du code du travail. Vous le savez, nous ne sommes pas tellement favorables à ces possibilités de dérogation qui engendrent, si elles ne sont pas encadrées par le principe de faveur, une fragilisation des droits des salariés. Ainsi, par ces dispositions nouvelles, la périodicité de l'obligation de négociation peut être modifiée pour passer d'une obligation annuelle à une obligation triennale, et ce sur tous les sujets des négociations prévues à l'article L. 2242-1

-et la qualité de vie au travail. Il ne s'agit donc pas de sujets mineurs. En supprimant l'article L. 2242-20, nous faisons disparaître toute possibilité de revenir, dans l'accord d'entreprise, sur la périodicité de ce type de négociations dont nous estimons qu'elles doivent se dérouler chaque année, dans l'intérêt des salariés. Tel est le sens de cet amendement 2016, est bien encadrée : elle suppose l'accord des partenaires sociaux dans l'entreprise et la signature d'un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, d'un plan d'action. Par ailleurs, toute organisation signataire d'un accord modifiant la périodicité de la négociation sur les salaires

et de l'employeur et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet outil permettra de mettre l'accent sur les problématiques essentielles qui doivent être traitées annuellement, tandis que les thématiques secondaires, ou plus consensuelles, pourront voir leur périodicité décalée.

doivent être triennales. Vous disiez, monsieur le rapporteur, que les thèmes importants vont pouvoir être débattus selon la volonté

ou s'accordent des augmentations, alors que leurs entreprises sont en difficulté, certains lorsque l'entreprise commence à licencier, d'autres lorsqu'ils demandent à leurs salariés de baisser de baisser leur salaire pour essayer de sauver l'entreprise, en se gardant bien, eux, de s'appliquer les mêmes règles. L'article L. 2254-2 du code du travail que « Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail. et de durée du travail. [ ...] L'accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : les dirigeants salariés aux autres salariés : les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.

avec peu de lustre et peu de réussite au niveau de la population. Les profits scandaleux existaient déjà. Ne venez pas reprocher à ceux qui sont au pouvoir depuis un mois de ne pas avoir fait ce que vous n'avez pas fait durant cinq ans

Il convient de trouver un équilibre dans le régime juridique de l'APDE afin de donner de la souplesse à l'entreprise, sans apparaître comme un repoussoir pour les syndicats et les salariés. Je crois que les règles actuelles sont équilibrées,

diminuer l'APL, à ponctionner les retraités, à mettre en place une politique complètement antisociale, alors que les inégalités sont la cause de la croissance molle

sur l'idée que chacun doit contribuer aux dépenses de la Nation par un effort non pas proportionnel mais progressif. Parce qu'il est progressif, il est progressiste ! Si j'ai bien compris, madame la ministre, monsieur le rapporteur, vous souhaitez promouvoir un dialogue progressiste

vont d'ailleurs à haute dose, et même à marche forcée : le Conseil d'État lui-même note que ce projet de loi d'habilitation « ne réserve pas la possibilité

véritable marche arrière : c'est seulement à partir de 1981 que la question de la négociation et de la présence syndicale dans l'entreprise a été inscrite dans la loi.

supprimé les alinéas 4 et 5, qui étaient importants en termes d'information et de représentation des salariés dans les conseils d'administration -ne me paraît pas renforcer le dialogue social. Tel est pourtant l'intitulé du projet de loi

ont rarement pour ambition principale de s'enrichir au détriment des droits sociaux de leurs employés, qu'ils connaissent et respectent. Ils n'ont pas l'immoralité de certains grands patrons dont le seul objectif est parfois d'amasser des milliards au détriment des droits sociaux et de l'environnement. Songez à la Françafrique

alors que la médecine du travail n'a pas les moyens de suivre tous les salariés, dans un contexte où les maladies professionnelles reconnues sont de plus en plus nombreuses ? Je pense en particulier au burn-out, dont personne aujourd'hui ne connaît l'origine. Si nous déplorons tous, syndicats eux-mêmes y compris, le manque d'engagement et d'investissement des salariés et des Français dans les organisations syndicales, ce n'est pas en réduisant leur poids dans le dialogue social, donc leur intérêt, que vous les rendrez attractives, Comme l'a dit notre président de groupe, oui à la flexibilité, mais oui à la sécurité ! De la sécurité, je n'en vois pas ; des dangers, j'en vois. Pour ces raisons et pour d'autres, nous

les questions de santé au travail. J'ajoute que chacune de ces instances a une histoire et surtout une raison d'exister, permettant aux salariés d'une entreprise d'intervenir et de s'exprimer. Par exemple, les CHSCT ont un rôle irremplaçable pour vérifier que les lois et règlements qui ont un rapport avec la sécurité au travail et la santé Ils sont également, grâce à la loi de 2013, des lanceurs d'alerte dans le domaine de l'environnement. Leur droit d'enquêter en cas de risque grave avéré ou d'atteinte à la santé est aussi d'importance. Enfin, ils analysent les propositions de l'employeur en matière d'aménagement important par exemple les grilles horaires, dès lors qu'elles ont une incidence sur la santé et la sécurité des salariés. Comme l'écrivait Louis-Marie Barnier, sociologue du travail, « Les élus du CHSCT constituent d'une certaine manière la mauvaise conscience de l'employeur, lui rappelant sans cesse les conséquences de ses décisions sur les salariés. » Très bien ! Les lois Auroux de 1982 mettaient en avant le projet d'un salarié-citoyen. Quant au droit européen, il impose à l'employeur, par la directive de 1989, de prendre toute mesure pour préserver la santé physique et mentale des salariés. Et pourtant, je constate que certaines organisations patronales considèrent bon nombre de ces prérogatives comme exorbitantes. Ce contre-pouvoir que constituent les CHSCT dans le domaine de la santé, de la sécurité, de l'organisation du travail semble en effet les gêner.

serait une excellente avancée, qu'il ne faut pas dénaturer en prévoyant des exceptions ou expérimentations. À l'évidence, madame la ministre, si vous n'imposez pas cette création, elle ne se fera pas. Les débats en commission l'ont bien montré au sujet du CHSCT, et je ne doute pas que nos discussions en séance le confirmeront, comme nous venons d'en avoir un aperçu. L'enjeu est de relancer le dialogue social ; il n'est pas utile de multiplier les instances ou d'en faire vivre de nouvelles telles que les CPRI, Il faut simplifier pour que les interlocuteurs soient moins nombreux, mais dotés de compétences élargies et renforcées. La deuxième partie de l'article 2 prévoit la mise en oeuvre du chèque syndical et la valorisation des carrières des représentants du personnel. Pourquoi pas ? Mais cela me semble bien modeste pour qu'il soit possible de parler de « mesures renforçant le dialogue social ». Il faut revoir en profondeur le rôle et le fonctionnement des organisations syndicales. Il faut notamment revoir leur financement pour le clarifier. Il faut réévaluer l'opportunité de la contribution patronale au dialogue social : prélever une cotisation obligatoire pour financer les syndicats est perçu par certains comme un véritable racket. Un tel prélèvement n'incite pas les syndicats à faire des efforts pour trouver de nouveaux adhérents.

Madame la ministre, vous semblez regretter le faible taux de syndicalisation, et par conséquent le faible nombre de délégués syndicaux dans les TPE et PME.

La réalité est qu'en 2017 être syndiqué est encore mal vu par certains patrons ; le risque de répression syndicale, s'agissant de l'avancement de carrière, est bien réel. Le 13 juillet dernier, le Conseil économique, social et environnemental a rendu un rapport intitulé « Repérer, prévenir, lutter contre les discriminations syndicales ». Y sont recensés les tentatives de licenciement abusif, les sanctions disciplinaires injustifiées, les chantages à l'emploi, les harcèlements ou encore les humiliations que que subissent certains salariés syndiqués au sein de leur entreprise. Selon le baromètre du Défenseur des droits et de l'Organisation internationale du travail cité dans ce même rapport, 11 % des salariés du privé et 11 % des agents du secteur public estiment en avoir été victimes eux pensent avoir été les témoins de discriminations syndicales. Cela est grave : ces actes discriminatoires ont également « valeur d'avertissement pour les autres salariés que l'on cherche à dissuader de s'engager syndicalement », précise le rapport. De son côté, la CGT a recensé en 2015, en son sein, 165 cas de médiations et actions en justice liées à la discrimination et à la répression syndicales. Madame la ministre, ce n'est pas en autorisant les employeurs à passer outre les délégués syndicaux

l'utilisation à mauvais escient des nouvelles technologies ; les difficultés dans les relations de travail, notamment avec le supérieur hiérarchique, lorsque l'isolement réduit les temps d'échange aux seules consignes. Votre conclusion était alors sans appel sur le rôle fondamental des CHSCT et la nécessité de leur renforcement. Aujourd'hui encore, quant à moi, je partage votre vision d'alors : le premier des droits des salariés est l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité au travail des personnels de son entreprise. Et la fusion des instances représentatives ne peut conduire

Où donc est passée la praticienne de 2010, madame la ministre ? Je conçois qu'il soit pénible, pour les employeurs, d'être déclarés responsables par les tribunaux pour n'avoir pas pour n'avoir pas pris en compte la santé et la sécurité des salariés. Mais quand pensez-vous aux salariés blessés ou malades ? Les salariés ont des devoirs et des obligations

les salariés des plateformes classées Seveso se battent avec de trop maigres moyens pour prévenir et faire reconnaître le danger auquel ils et elles ont été exposés, leurs maladies professionnelles, les conséquences pour leurs familles. Je pense également, dans le secteur de l'énergie,

Madame la ministre, à lire votre projet de loi, on constate que le dialogue social que vous appelez de vos voeux est totalement asymétrique. Comment justifier que court-circuiter les syndicats, réduire le nombre d'instances et, de fait, le nombre d'élus, vivifierait la démocratie ? Au lieu de proposer des mesures contradictoires avec les objectifs annoncés, il conviendrait plutôt de s'interroger sur les raisons de la faible syndicalisation. Si les organisations syndicales doivent s'interroger sur leur modèle d'organisation, il faut aussi explorer d'autres pistes. D'une part- je ne ferai qu'évoquer ce point -, madame la ministre, vous vous doutez bien qu'il est plus difficile de s'engager lorsque la précarité et le risque de déclassement sont forts. D'autre part- j'insiste sur ce point -, la peur du chômage et le comportement trop souvent impuni d'employeurs peu amènes avec leurs salariés syndiqués ne peuvent que freiner l'engouement pour le syndicalisme. Poursuites judiciaires répétées jusqu'au dernier recours pour épuiser les salariés concernés, avancements freinés, brimades, délégitimation devant les collègues : tous les moyens sont bons, aux yeux de certains employeurs, pour affaiblir les contre-pouvoirs dans l'entreprise. On pourrait citer la SNCF, condamnée quatorze fois en 2015 après plusieurs années de procédures

Jacques Toubon, et comme le montre l'avis assorti de vingt-trois recommandations du CESE du 13 juillet dernier. Dans plus du tiers des entreprises interrogées par le ministère du travail, 45 % des représentants du personnel syndiqués déclarent que leur mandat a été un frein pour leur carrière, contre 4 % des représentants non syndiqués, alors même que le salaire de ces travailleurs est plus faible. Ces pratiques répressives et discriminatoires ont forcément des conséquences sur l'engagement des salariés entre 36 % et 40 % des salariés déclarent que le premier frein à la syndicalisation est la peur des représailles émanant de la direction de l'entreprise. Si le Gouvernement veut inciter à la syndicalisation, qu'il renforce la législation, qu'il fasse appliquer les lois existantes et qu'il lutte contre ces pratiques d'un autre temps ! À ce titre, le soutien quasiment sans faille des DIRECCTE à des licenciements bien souvent condamnés par la justice ne peut qu'interroger ! Entre 2010 et 2014, l'administration a accepté plus des trois quarts, près de 77 %, des demandes de licenciement,

loi ! Madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance au-delà de minuit et jusqu'à zéro heure trente afin de poursuivre l'examen de ce texte, et surtout de pouvoir discuter des amendements de suppression

sur l'article. Les personnes en situation de handicap ont trois fois moins de chances d'occuper un emploi et deux fois plus de risques de connaître le chômage. Seulement 43 % des personnes reconnues en situation de handicap sont actives, et 35 % sont en emploi. Le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à celui de la population générale. Les personnes en situation de handicap sont souvent moins qualifiées, moins formées et plus âgées que la population générale. Le nombre de personnes en situation de handicap qui travaillent augmente. Aujourd'hui, près de 1 million de personnes handicapées travaillent, dont 80 % en milieu ordinaire de travail. Quand elles travaillent, les personnes en situation de handicap occupent plus souvent un emploi peu ou pas qualifié, plus souvent que d'autres à temps partiel ou en situation de sous-emploi. Le handicap est la deuxième cause de discrimination recensée par le Défenseur des droits, et ce principalement dans l'emploi. Les personnes en situation de handicap ont des qualités, des capacités et des compétences qui doivent pouvoir s'exprimer sur le marché du travail. Dans le soutien à la politique inclusive des personnes handicapées voulue par le Président de la République, au regard de cette situation, la commission travail-emploi-formation du Conseil national consultatif des personnes handicapées, que j'ai l'honneur de présider, recommande, d'une part, de ne pas dissocier les questions relatives à l'emploi des personnes en situation de handicap de celles qui sont liées à la rénovation de notre modèle social d'assurer une sécurisation des parcours vers et dans l'emploi pour tous. Par conséquent, je demande que le Gouvernement mène systématiquement des études d'impact des réformes envisagées sur l'emploi des personnes en situation de handicap et des proches aidants aidants en matière tant d'accès, d'évolution professionnelle que de maintien dans l'emploi, afin de généraliser et de rendre habituelle l'obligation de recrutement de 6 % de personnes handicapées dans les effectifs salariés des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.

La fusion doit permettre de simplifier le dialogue social, mais aussi d'en renforcer le contenu stratégique. La représentation des salariés est aujourd'hui morcelée en quatre instances différentes au sein de l'entreprise : délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et délégués syndicaux.

Le système est chronophage, complexe et, en partie, inefficace. Il aboutit à un dialogue social éclaté et à des complications du travail supplémentaires. La quasi-totalité des pays qui entretiennent un dialogue social très développé ont moins d'instances que nous.

L'ensemble des compétences du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du CHSCT doivent être transférées au nouveau comité. Il ne doit surtout pas être question de baisser la garde sur la santé et la sécurité au travail. À cet égard, je suis favorable à la constitution d'une commission spécifique. La présence d'une instance bénéficiant de la vision stratégique globale ne fait pas obstacle à la création d'une commission spécialisée travaillant sur les métiers dangereux. Un amendement a été déposé en ce sens. Enfin, et c'est essentiel, la compétence d'ester en justice doit être transférée à cette nouvelle instance. J'insiste sur un dernier point de vigilance. Puisqu'il est également prévu de limiter le nombre de mandats des représentants du personnel, il est important d'envisager un encadrement du retour à l'emploi des salariés protégés, afin d'éviter la chasse aux sorcières qui a parfois lieu et est source d'un nombre non négligeable de contentieux prud'homaux.

Dans certains cas, en fonction des secteurs d'activité ou des effectifs, il pourrait être envisagé de regrouper à moyens constants les compétences du comité d'entreprise et du CHSCT dans une instance unique, sous réserve de l'accord des partenaires sociaux.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les prises de parole sur l'article. Nous examinerons les trois amendements tendant